Madame la ministre, mes chers collègues, je suis particulièrement heureux de saluer la présence dans la tribune d'honneur de M. Thomas Hefti, président du Conseil des États de la Confédération helvétique, de M. Charles Juillard, président du groupe d'amitié Suisse-France, et de Mme Simone de Montmollin, conseillère nationale, vice-présidente de la délégation pour les relations avec le Parlement français. Ils sont accompagnés par notre collègue Bernard Bonne, président du groupe d'amitié français entretient depuis toujours d'excellentes relations de confiance et d'amitié avec l'Assemblée fédérale suisse. La présence de nos collègues dans l'hémicycle aujourd'hui l'illustre parfaitement, tout comme la visite en octobre 2021

nos pensions de retraite devraient baisser de 8 % car l'équilibre que nous avons construit avec les efforts de tous les médecins, actifs et retraités, serait rompu et ce ne serait pas acceptable.

Le Gouvernement peut décider de défiscaliser les médecins pour les inciter à poursuivre leur activité, mais la sécurité sociale n'a pas à supporter de nouvelles pertes de recettes.

Toutefois, je voterai contre cet amendement : ce que proposent le Gouvernement et la commission me paraît aller dans le bon sens.

madame la ministre, je voudrais vraiment abonder dans le sens de la question qui vous a été posée. Y a-t-il possibilité d'une compensation pour la caisse qui ne va pas percevoir ces cotisations ?

ils font ce qu'ils veulent. Vous allez les inciter à prendre leur retraite plus tôt, tout en nourrissant un phénomène d'exonération générale de cotisations sans droits ouverts derrière.

on va leur permettre de prendre la retraite, mais, au premier jour de leur retraite, de pouvoir continuer leur activité et de garder tous les revenus qui sont les leurs, pour eux, sans payer de cotisations retraite nouvelles. Tous les territoires de France connaissent une pénurie de médecins. Si la suppression du doit apporter une réponse à cet état de fait, ses effets ne seront effectifs que dans plusieurs années seulement. D'ici là, il est important de maintenir en activité les médecins actuellement en place, et ce le plus longtemps possible. En Île-de-France, premier désert médical en France avec plus de 96 % du territoire considéré comme une zone d'accès aux soins difficile, soins difficile, près de la moitié des médecins libéraux en activité ont plus de 60 ans, et un quart d'entre eux a plus de 65 ans. Dans ce contexte, il est tout à fait anormal que les médecins libéraux en cumul emploi-retraite continuent à payer des cotisations retraite retraite ne leur ouvrant aucun droit supplémentaire. Cela représente en moyenne 9 850 euros de cotisation annuelle pour un médecin en secteur 1 et 16 443 euros pour un médecin forte désincitation à la poursuite de leur activité. Pour encourager les médecins libéraux à rester en activité et même faire revenir certains retraités, il paraît nécessaire de supprimer cette cotisation pour les médecins en cumul emploi-retraite. La mesure a déjà fait ses preuves

ramenant le taux de cotisations des professionnels de santé libéraux affiliés au régime des PAMC (praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés), soit 9,81 %, à hauteur du taux appliqué au RSI (régime de la sécurité sociale) pour 2016 a également introduit une taxe additionnelle de 3,25 % applicable aux revenus tirés d'une activité non conventionnée ou des dépassements d'honoraires pour les seuls professionnels de santé affiliés au régime des PAMC. Cette taxe s'applique ainsi à des revenus tirés d'activités de soins, selon les termes de la convention négociée avec l'assurance maladie, ou contribuant au bon fonctionnement et à l'amélioration du système de santé. La suppression de cette taxe additionnelle répond plus largement à un souci d'équité à l'égard des autres professions libérales et indépendantes auxquelles cette taxe n'est pas applicable, pour les activités ci-dessus mentionnées. Elle vise à mettre un terme à cette discrimination entre professionnels de santé libéraux selon leur régime d'affiliation et répond à la politique gouvernementale d'harmonisation des cotisations sur les revenus d'activité.

Il s'agissait en effet de maintenir le niveau de cotisation des médecins pratiquant des dépassements d'honoraires, de façon à produire un effet désincitatif.

à se désaffilier du régime des praticiens et auxiliaires médicaux, de façon à ne pas être redevables de cette contribution. L'article 49 tend d'ailleurs à étendre cette faculté. Dans ces conditions, je demande le retrait de ces amendements

de santé de 2016 devait garantir un meilleur accès aux soins, en incitant les praticiens au respect des tarifs conventionnels et à la limitation des dépassements d'honoraires. Cette contribution additionnelle n'est applicable qu'aux seuls dépassements d'honoraires et revenus non conventionnés. C'est une contrepartie à la participation financière de l'assurance maladie au paiement des cotisations sociales dues par ces praticiens au titre de leurs revenus conventionnés. La cette contribution ira à l'encontre, je crois, des objectifs d'accès aux soins et de régulation des tarifs pratiqués par les professionnels de santé.

d'une exonération de l'ensemble des cotisations pendant quatre ans. Je préfère que nous attendions la réforme des retraites pour en discuter et prendre les mesures qui s'imposent dans ces territoires,

M. Christian Klinger. Cet amendement a pour objet de simplifier les procédures de déclaration d'emplois ponctuels, pour les petites associations, dans le cadre de manifestations de bienfaisance ou de soutien qu'elles organisent à leur profit exclusivement. Pour organiser ces manifestations, il est souvent fait appel à des bénévoles et, en cas de manque de bénévoles, à des emplois ponctuels, le plus souvent pour quelques heures seulement, pour sécuriser des parkings ou tenir les toilettes par exemple. Aujourd'hui, l'Urssaf impose aux représentants des associations de réaliser des déclarations pour chacun de ces emplois, même pour quelques heures de poste, alors qu'ils répondent aux critères de réduction générale des cotisations patronales sur les bas salaires. « le chèque emploi associatif a été mis en place sur le modèle du Cesu et, en théorie, il permettrait aux associations, même aux plus petites d'entre elles, de recruter des personnes pour une courte durée pour un événement particulier. Mais, dans les faits, les représentants des associations en font peu l'usage. Dans un souci de simplification, cet amendement vise à exclure de la liste de l'assiette de la contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement ces emplois ponctuels, uniquement au bénéfice des associations et des fondations, ainsi que des organismes permanents à caractère social des collectivités locales et des entreprises, et ce dans la limite de six manifestations par an.

organisées dans l'année à leur profit exclusif par les organismes désignés ». Il suffit de transposer la dérogation en matière de TVA, pour faire en sorte que la règle sociale soit la même

libre et gratuite, les salariés que vous mentionnez sont quant à eux, rappelons-le, liés aux associations par un contrat de travail. Ils sont rémunérés au titre de l'activité pour laquelle ils ont été recrutés. Les rémunérations qui leur sont versées entrent dans l'assiette de la CSG telle que définie par le code de la sécurité sociale. Une exclusion de l'assiette de la CSG et, par conséquent, de cotisations sociales pour ces rémunérations aurait pour effet de créer une différence de traitement manifeste à l'égard des autres salariés, pour des revenus et des situations identiques. Elle serait aussi possiblement contraire au principe d'égalité devant les charges publiques.

de l'obligation de réaliser les formalités déclaratives que vous mentionnez et qui sont indispensables à l'ouverture de droits sociaux de ces salariés, notamment en cas de maladie, de chômage ou pour leur future retraite.

Aujourd'hui, ces gens-là sont payés en liquide, pris sur la caisse de la recette de la journée de l'activité de la manifestation annuelle, ce qui leur permet de survivre et de payer leurs quelques frais. Je ne parle pas des employés qui sont salariés à titre habituel. Il s'agit vraiment

Vous l'écrivez vous-même, non sans talent, si vous me permettez, monsieur le sénateur, « le chèque emploi associatif a été mis en place sur le modèle du Cesu et, en théorie,

on est bien content de se tourner vers la sécurité sociale, qui prend en charge les différents soins. Plutôt que de chercher à faire des économies sur la sécurité sociale, pourquoi ne pas demander l'exonération des droits d'auteur ? C'est une boutade, mes

offrant aux salariés économiquement fragiles une couverture supplémentaire. Complémentaires des assurances obligatoires, ces produits d'assurance sont pris en charge à 100 % par l'entreprise.

Afin de protéger le pouvoir d'achat des salariés, cet amendement vise à exclure de la qualification d'« avantage en nature » la prise en charge par l'employeur du coût des contrats d'assurance de ce type. Il me semble que cette proposition s'inscrit dans le prolongement du texte que nous avons voté pour protéger le pouvoir d'achat.

? J'ajouterai à ce que vient de dire Mme la rapporteure générale que la fourniture ou la mise à disposition d'un bien ou d'un service qui permet au salarié de faire l'économie de frais qu'il aurait dû normalement supporter, c'est la définition même d'un avantage en nature, qui constitue et bien une forme de rémunération du salarié. C'est pour cette raison qu'il est clairement précisé dans le code de la sécurité sociale que tout avantage en nature doit être,

de sécurité sociale, mais aussi- nous ne cessons d'en parler cet après-midi -pour garantir l'acquisition de droits sociaux par le salarié. De surcroît, une telle exonération créerait une iniquité de traitement entre des salariés qui perçoivent une rémunération totale identique selon que celle-ci est versée intégralement sous forme de salaire

fois la valeur du plafond annuel de la sécurité sociale, soit dans la limite de 164 544 euros brut annuels pour 2020, mais à une fois ce même plafond. À l'heure actuelle, cet abattement profite mécaniquement aux revenus aisés. Nous proposons d'en abaisser le plafond

par des non-résidents sont assujettis à divers prélèvements sociaux dont le taux est, depuis le 1 janvier 2017, de 17,2 %, alors même que ceux-ci ne bénéficient en contrepartie d'aucune prestation sociale. Cette imposition a été jugée incompatible avec le principe d'unicité de la législation de sécurité sociale consacré par le règlement (CE) n° 883/2004. La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a ainsi considéré que les personnes affiliées à un régime de sécurité sociale d'un État membre de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse ne peuvent être assujetties en France à des prélèvements sociaux sur leurs revenus fonciers. notre droit en conformité avec le droit européen, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 a exonéré de la CSG-CRDS les non-résidents affiliés à un système de sécurité sociale de l'Union européenne, de l'Espace économique européen et de la Suisse. En revanche, l'assujettissement aux prélèvements sociaux des non-résidents d'un État tiers assujettissement constitue une iniquité de traitement fiscal, une réelle discrimination face à l'impôt ; en outre, il décourage l'investissement immobilier en France de nos compatriotes établis à l'étranger. Les non-résidents s'acquittent dans la majorité des cas, en plus de la CSG-CRDS due en France, d'une cotisation soit à une caisse de sécurité sociale à adhésion volontaire telle que la Caisse des Français de l'étranger (CFE), soit au système de protection sociale de leur pays de résidence. Ainsi subissent-ils une double imposition finalité sociale. Au nom du principe d'équité fiscale, l'exonération de CSG-CRDS devrait être généralisée à tous les non-résidents, où qu'ils habitent. L'amendement

entre les Français affiliés à un régime de sécurité sociale d'un pays de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen (EEE), d'une part, et les Français affiliés à un régime de sécurité sociale d'un pays situé hors de l'Union et de l'EEE. Cet amendement a déjà été adopté

physiques (IRPP) en France à raison de certains de leurs revenus et simultanément assujettis à quelque titre que ce soit à un régime obligatoire français d'assurance maladie. Le présent amendement tend à reprendre cette solution.

sont affiliés à un régime obligatoire de protection sociale, la caisse de prévoyance sociale, et leur domicile fiscal n'est pas en France ; pourtant, ils ne sont pas exonérés de CSG-CRDS et sont ainsi soumis à une double imposition. Cette inégalité de traitement est d'autant plus importante que la loi du 3 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 a bien prévu une exonération de ces prélèvements pour les Français résidents au sein de l'Espace économique européen et en Suisse. Les articles I et VI de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen posent le principe d'égalité devant la loi fiscale, en vertu duquel le même régime fiscal doit s'appliquer à tout contribuable placé dans une situation identique. Par ailleurs, la Polynésie française et l'État ont signé en 1957 une convention fiscale tendant à éliminer les doubles impositions et à établir des règles d'assistance mutuelle administrative pour les impositions des revenus des capitaux mobiliers. Or celle-ci ne couvre ni la CSG ni la CRDS, ces cotisations sociales n'ayant été respectivement créées

À la suite de plusieurs arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne, les arrêts et, le Gouvernement a été contraint de proposer au Parlement l'exonération de ces prélèvements en faveur de nos compatriotes assurés dans l'Union européenne. L'article 26 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 a acté une telle modification. Mais cette réforme bienvenue a laissé sur le carreau nos compatriotes domiciliés hors de l'Union. Cette loi a donc créé une discrimination de fait entre les Français de l'étranger selon leur lieu de résidence et leur régime d'affiliation.

sociale, même minimale, ils contribuent en effet au financement de régimes obligatoires de sécurité sociale, d'assurances privées coûteuses ou du régime volontaire de la CFE

Le Conseil constitutionnel n'a pas davantage trouvé à redire sur cette différence entre non-résidents communautaires et non-résidents non communautaires. La législation française est donc parfaitement en phase avec la jurisprudence constitutionnelle et communautaire. Selon ces hautes juridictions,

Le fait que ces contributions servent à financer des régimes sociaux ne change rien à l'affaire : tous les Français, riches ou modestes, acquittent la CSG et la CRDS sur leurs revenus d'épargne sans que cela leur crée le moindre droit social. fond, contester cet assujettissement reviendrait à revendiquer aussi que ces revenus financiers français ne soient pas soumis non plus aux impôts d'État, comme l'impôt sur le revenu ou les prélèvements de solidarité, au prétexte que les non-résidents utilisent moins les routes ou les écoles françaises que les autres J'ajoute que la plupart de ces amendements visent non pas seulement nos compatriotes établis hors de France, mais également les revenus financiers de source française d'étrangers parfois fortunés. Notre priorité est-elle vraiment de tels revenus de CSG et de CRDS ? dont les auteurs ont tâché d'échapper à cette dernière critique, je ne pense pas que le Conseil constitutionnel considérerait qu'il est possible de réserver une exonération de CSG ou de CRDS aux non-résidents ayant été assurés sociaux en France pendant au moins cinq ans. La différence de situation entre ces non-résidents et les autres non-résidents ne semble pas justifier une telle différence de traitement fiscal. Il en est d'ailleurs de même pour les assurés au régime de la Polynésie française.

puisqu'on parle non plus de cotisation mais d'impôt, à une rupture d'égalité devant l'impôt.

nous considérons que la rupture d'égalité devant l'impôt peut être autorisée, puisqu'une partie des Français seulement, ceux qui vivent dans l'Union européenne, sont exonérés

Cet amendement de bon sens vise à aligner le taux de CSG applicable aux revenus du capital sur celui des revenus d'activité. En 2018, le Gouvernement a relevé de 1,7 point la CSG sur les revenus d'activité et de remplacement sur les salaires et les pensions de retraite, tandis que la CSG sur les revenus du capital n'a progressé que de 1 point. En 2022, les dividendes versés par les entreprises du CAC 40 ont battu des records, pour atteindre 44,3 milliards d'euros. Cet amendement de repli, vous l'aurez compris, est une mesure de justice

est à M. Jean-Jacques Michau. Par cet amendement, il est proposé d'augmenter de 0,25 point la CSG sur les revenus du capital- produits de placement et patrimoine -, afin de dégager des recettes supplémentaires pour la sécurité sociale.

le report, voire l'abandon, d'une loi Grand Âge et autonomie, autrement dit le renoncement à trouver des financements supplémentaires à la hauteur des défis du vieillissement, est incompréhensible. Or, pour 2023, le texte ne prévoit que 3 000 équivalents temps plein (ETP) dans les Ehpad, loin des 50 000 annoncés d'ici à la fin du mandat. Cela représente moins d'un demi-poste par établissement. L'argument présenté selon lequel les grandes difficultés de recrutement des établissements justifient le très faible nombre de créations de postes pour cette année n'est pas valable. Cet amendement vise à dégager environ 250 millions d'euros afin de financer 4 500 ETP supplémentaires. Cela représenterait ainsi 7 500 postes, soit au moins 1 ETP par établissement. Il s'agit là du minimum, car les besoins sont évidemment bien plus importants. Cet amendement tend à accélérer la trajectoire annoncée.

à ne pas augmenter le niveau de la fiscalité. J'ajoute que la CSG sur les revenus du capital est passée à 9,2 % en 2020, sans oublier la CRDS au taux de 0,5 %, le prélèvement de solidarité attribuée à l'État depuis 2018 au taux de 7,5 points, ce qui porte à 17,2 % le niveau des prélèvements sociaux sur le capital, auxquels s'ajoute un taux de 12,8 % au titre de l'impôt sur le revenu, soit un total

en matière d'investissements directs en France, notamment de nos voisins européens, nous demeurons la première place en matière d'attractivité. L'investissement des entreprises, dont j'ai l'honneur d'être chargée, a résisté sur l'année

vise à alléger la fiscalité sur les véhicules mis à la disposition permanente des intervenants à domicile par leur employeur afin d'effectuer leurs tournées au domicile, notamment des personnes âgées en perte d'autonomie ou en situation de handicap, dans le but d'accroître l'attractivité des métiers du domicile, particulièrement en tension. Le secteur de l'aide à domicile est confronté à d'importantes difficultés de recrutement. Parmi ces difficultés figure le fait que le personnel ne disposant pas de véhicule n'est que peu employable dans ce secteur. En l'état actuel du droit, seule la mise à disposition d'un véhicule à un salarié pour un usage exclusivement professionnel n'est pas soumise à charges sociales. Le salarié doit rapporter le véhicule de service, chaque soir, à l'entreprise., l'utilisation exclusive à titre privatif d'un véhicule mis à la disposition du salarié de façon permanente constitue un avantage en nature. En effet, lorsqu'un employeur met à la disposition permanente d'un salarié un véhicule dont il est propriétaire ou locataire, l'utilisation privée qui en est faite représente un avantage en nature soumis à cotisations et, en conséquence, considéré comme un revenu imposable pour le salarié. Cet amendement vise à exclure des bases de cotisations de sécurité sociale et, partant, de la base de revenu imposable les véhicules mis à disposition par les structures d'aide à domicile à leurs salariés sans distinction des périodes d'utilisation professionnelle et non professionnelle. Cette mesure permettrait d'améliorer le pouvoir d'achat de ces salariés de première ligne et d'augmenter grandement leur employabilité, sans grever les budgets des services d'aide à domicile.

: la mise à disposition d'un véhicule pour un usage professionnel ne constitue pas un avantage en nature, à la différence d'une mise à disposition d'un véhicule pour un usage personnel.

: La parole est à Mme Sylvie Vermeillet. En soutien au pouvoir d'achat, certaines entreprises et collectivités volontaires accompagnent, sous conditions de ressources et d'éloignement géographique du lieu de travail, les salariés dépendants de leur voiture pour effectuer leur trajet domicile-travail en les faisant bénéficier d'un chèque carburant cofinancé par les deux entités. Compte tenu des importantes tensions inflationnistes qui perdurent, cet amendement vise à faciliter cette démarche jusqu'à la fin de l'année 2023.

pour leurs déplacements professionnels domicile-travail, à 500 euros par an, ce qui permet aux salariés de bénéficier d'une aide de 50 euros par mois. Mis en place, notamment, par le conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, ainsi que par d'autres régions, ce dispositif volontaire accompagne les salariés dans leur trajet de travail sans aucun coût de gestion : il consiste en un simple paramétrage du logiciel de paie de l'entreprise. Il ne coûte rien à l'État ; il est validé et encouragé par les partenaires sociaux, de la CGT au Medef,

Mme Pascale Gruny. Cet amendement a pour objet d'assimiler clairement et de manière pérenne l'indemnité complémentaire d'activité partielle à un revenu de remplacement. Compte tenu du contexte lié à l'épidémie de covid-19, l'article 8 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 prévoyait, pour les années 2021 et 2022, un régime dérogatoire en vertu duquel les indemnités complémentaires versées par l'employeur dans la limite de 3,15 Smic sont assujetties au régime social applicable aux revenus de remplacement. Ce dispositif parvenant à échéance au 31 décembre 2022, le site Urssaf précise qu'à compter de 2023 l'indemnité complémentaire versée par l'employeur devra être assujettie aux cotisations et contributions sociales applicables aux revenus d'activité dans dans son intégralité. La mesure proposée semble d'autant plus justifiée que, en l'absence de doctrine clairement établie à ce sujet, de nombreuses entreprises ont conclu des accords basés sur l'interprétation fournie par la circulaire de la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle du 12 juillet 2013 relative à la mise en oeuvre de l'activité partielle, laquelle assimile explicitement la complémentaire versée par l'employeur dans le cadre d'un accord de branche, d'entreprise ou d'une décision unilatérale d'entreprise à un revenu de remplacement. Quel

Vous proposez, madame la sénatrice Gruny, de pérenniser un régime social provisoire, qui a été appliqué aux indemnités complémentaires versées aux salariés placés en activité partielle pendant la crise covid. Compte tenu du recours accru au dispositif d'activité partielle lors de la crise sanitaire, le traitement social favorable des indemnités légales d'activité partielle a été étendu, à titre dérogatoire, aux indemnités complémentaires. Ainsi, depuis le 1 janvier 2021 et jusqu'au 31 décembre de cette année, les indemnités complémentaires d'activité partielle sont exonérées de cotisations sociales et assujetties au taux de 6,2 points de CSG et de 0,5 point de CRDS. Toutefois leur fraction qui excède 3,15 Smic est assujettie aux cotisations sociales comme des revenus d'activité normaux. Vous justifiez votre amendement par le fait que certaines entreprises ont déjà conclu des accords sur la base de la doctrine établie par la circulaire du 12 juillet 2013, qui assimilerait ces indemnités à des revenus de remplacement. Toutefois, la circulaire indique également que l'exclusion d'assiette sociale des indemnités d'activité partielle ne valait que dans la limite des taux de remplacement prévus au sein du code du travail. Depuis lors, les dispositions de la LFSS pour 2021 ont clarifié la situation, prévu un terme au régime social dérogatoire admis pendant la crise et laissé un temps suffisant aux employeurs ainsi que de la visibilité pour se préparer à un retour au régime pérenne, cohérent avec le droit commun. Considérer ces indemnités comme des revenus de remplacement, ce qui est inexact, serait donc injustifié

La troisième loi de finances rectificative pour 2020 du 30 juillet 2020 a prévu, pour les exploitants agricoles ayant subi des pertes importantes pendant la période de confinement, la possibilité d'opter pour le calcul des cotisations dues au titre de 2020 sur le revenu professionnel de l'année 2020. Toutefois, pour de nombreux exploitants, les pertes résultant de la crise sanitaire seront constatées dans les bilans clos en 2021, notamment dans le cas où l'exercice ne coïncide pas avec l'année civile. Ainsi, pour avoir un effet, l'option pour le calcul des cotisations sociales sur les revenus de l'année doit aussi pouvoir s'appliquer en 2021. À défaut, l'exploitant dont dont le bilan clos dans les premiers mois de l'année 2020 reflète davantage l'activité de l'année 2019 et dont la baisse d'activité subie en 2020 sera répercutée sur le bilan clos en 2021 se verrait appeler, en 2021, des cotisations sociales calculées sur la base du revenu de l'activité d'avant-crise, ce qui serait très difficile à supporter. Asseoir les cotisations sur les revenus contemporains est donc le meilleur système pour adapter leur montant aux capacités réelles des exploitants et pour tenir compte de la grande hétérogénéité des impacts économiques du covid-19 en agriculture. Quel ? Cher collègue, vous souhaitez la prolongation sur l'année 2021 d'un dispositif dérogatoire de calcul des cotisations sociales pour les exploitants agricoles touchés tant par les intempéries que par les conséquences de la crise épidémique de covid-19.

à distribuer les produits du tabac dans le cadre d'un contrat de gérance passé avec l'État, qui en fait des préposés de l'administration. Depuis 2018, les buralistes se sont engagés dans une grande démarche de transformation de leurs points de vente ainsi que de leur modèle économique, ce qui fait d'eux des commerçants d'utilité locale à part entière et non plus de simples débitants de tabac. Ils se retrouvent, malgré tout, confrontés depuis plusieurs années à l'essor du marché parallèle du tabac- contrebande, contrefaçon, achats transfrontaliers. À la suite du confinement, on a pu mesurer que plus de 30 % des cigarettes consommées en France étaient achetées en dehors du réseau des buralistes, lesquels sont pourtant les seuls habilités par l'État à vendre ces produits. L'introduction par cet article de nouvelles dispositions fiscales conduisant à augmenter les prix des produits du tabac renforcera mécaniquement ce marché parallèle et les multiples effets néfastes qu'il engendre. Les points de vente à la sauvette, déjà si nombreux, sont ainsi appelés à se multiplier, tandis que la contrefaçon de cigarettes se renforcera. Au mois de septembre dernier, une nouvelle usine de contrefaçon a été découverte en Seine-et-Marne- c'est la deuxième en moins d'un an. Une telle révision de la fiscalité risquerait aussi de précipiter massivement de nouveaux consommateurs de tabac vers ce marché parallèle, de plus en plus capté par les mafias qui organisent ces trafics.

risque de grever considérablement la situation financière déjà précaire des consommateurs. Il serait au contraire bien plus opportun de mettre l'accent sur la prévention du tabagisme, tout en continuant à soutenir le réseau des buralistes, dont la réactivité et le dévouement pendant la crise sanitaire ne sont plus à démontrer. Ces véritables commerçants d'utilité locale tiennent bien souvent le dernier commerce présent dans nos villages et nos quartiers. Cette mesure comporte de nombreux effets pervers et risque de se révéler totalement inefficace, voire contre-productive.

une indexation sur l'inflation sans plafonnement, afin d'éviter une baisse du prix relatif du tabac qui affaiblirait les résultats engrangés ces dernières années. Si cette indexation n'était pas réalisée, tous les efforts engagés depuis 2017 seraient annulés au regard du prix relatif des tabacs

La nouvelle rédaction introduite par le Gouvernement a conservé plusieurs principes importants, que nous approuvons, comme l'accélération et le déplafonnement de la prise en compte de l'inflation pour le calcul de l'accise sur les produits du tabac.

à la définition très restrictive, d'autre part, en allégeant la fiscalité applicable à ces produits par rapport à la proposition initiale, surtout pour ce qui concerne les « autres tabacs à chauffer ». Il est donc préférable de s'en tenir aux modifications proposées par cet article dans sa version d'origine.

L'industrie du tabac ne manque pas d'imagination lorsqu'il s'agit de protéger ses parts de marché. Je crois qu'il faut s'en tenir à une rédaction stricte concernant la fiscalité de tous ces produits, dont le tabac à chauffer. Nous souhaitons donc revenir à la version initiale de l'article 8, qui allait plus loin que la version actuelle, en taxant plus fermement le tabac chauffé, dont les conséquences pour la santé sont tout aussi délétères, contrairement à ce que l'industrie laisse entendre. La taxation à l'unité est plus adaptée que la taxation au poids, lequel peut être diminué par l'industrie dans une stratégie d'évitement fiscal.

projet de loi de financement de la sécurité sociale était une occasion de veiller à ce qu'il n'y ait pas de rupture dans les politiques menées depuis désormais bien longtemps- et c'est heureux -pour réduire la consommation de tabac dans notre pays.

souligne toutefois, l'expérience montre que l'utilisation du poids du tabac comme base de taxation encourage l'industrie à produire des cigarettes plus légères, mais non moins nocives,

de renforcer ainsi les recettes fiscales étatiques, le Gouvernement tente de justifier l'augmentation de la fiscalité par un souci de prévention en matière de santé publique. Pourtant, cette nouvelle augmentation conduirait irrémédiablement à un report de la consommation vers des produits contrefaits, au détriment de la santé des consommateurs, des buralistes et des finances publiques, surtout dans ces proportions. J'en parle en connaissance de cause, puisque l'État

la Première ministre elle-même a déclaré que, dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale, l'augmentation de la fiscalité devait être alignée sur le taux de l'inflation. Pour ces raisons,

Ce nouveau dispositif créait dès lors une augmentation totale de 7,10 % des prix du tabac. Le texte sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité a évolué partiellement, afin de limiter le développement du marché parallèle. Le dispositif proposé reste cependant inchangé en ce qui concerne les autres catégories

vers le marché parallèle et, tout particulièrement, vers la contrefaçon et la contrebande. Le texte soumis au Sénat prévoit toujours une hausse de plus de 7,1 % de la fiscalité applicable aux cigarettes et une hausse de plus de 9 % pour le tabac à rouler.

de compromis vise donc à indexer et à plafonner le tarif et le minimum de perception des trois principales catégories des produits du tabac sur l'inflation prévue sur la seule année 2022, et non sur le cumul des deux années 2021 et 2022.

et l'allégement de la fiscalité prévue pour l'ensemble de ces produits, notamment les autres tabacs à chauffer, pourraient inciter les producteurs à effectuer de légères modifications de longueur, de diamètre ou de composition de leurs produits pour basculer

Par conséquent, je serai, au nom du Gouvernement, défavorable à l'ensemble des amendements et des sous-amendements.

que l'engagement pris par Olivier Dussopt soit mis à mal, puisque nous sommes en train de légiférer pour 2023. Je mets aux voix

dans la mesure où de nouveaux produits nicotinés ont émergé depuis quelques années. Ce phénomène est la conséquence directe de la hausse constante de la fiscalité des cigarettes et de la volonté des industriels d'inventer de nouveaux moyens de consommation de la nicotine : le vapotage et le tabac à chauffer, qui sont les premières traductions de cette évolution des mentalités et des pratiques, mais pas seulement ! Aujourd'hui, il y a également ce qu'on appelle le , ce tabac humide en sachet qu'on place entre la gencive et la lèvre. la lèvre. Des produits autres que ceux que nous avons préalablement mentionnés et qui ne constituent pas des substituts nicotiniques pour cesser de consommer du tabac sont d'ores et déjà sur le marché français. Leur consommation est à l'heure actuelle résiduelle, ce qui explique une certaine méconnaissance. Il est question ici de les réglementer en matière fiscale, en adéquation avec la réglementation de plusieurs États de l'Union européenne. En effet, la majeure partie des pays ont déjà décidé de les inscrire dans leurs systèmes fiscaux nationaux et ont mis en place une taxation au poids, comme l'Italie. Cet amendement vise donc à harmoniser le mode de calcul des taxes entre les pays européens, dans un objectif de santé publique.

Comment expliquer en effet, alors que près d'un quart des Français font une consommation excessive d'alcool, que les prix des boissons alcoolisées ne suivent pas la même progression que les biens de consommation courante et apparaissent ainsi relativement moins chers ?

C'est pourquoi elle a émis un avis favorable sur la proposition de taxe sur les , ces cigarettes électroniques jetables dont le succès chez les jeunes est rapide, voire inquiétant si l'on tient compte de ce que dit le Haut Conseil de la santé publique sur la responsabilité du vapotage dans l'entrée dans le tabagisme. La commission a, pour la même raison, approuvé un amendement visant à créer une taxe sur les bières aromatisées sucrées ou édulcorées, très prisées du jeune public, taxe dont le mécanisme ne toucherait pas les petites brasseries- je le dis à l'attention de mes collègues de l'est de la France.

Troisième principe qui a guidé nos débats : la prudence dans le recours à l'outil fiscal pour certaines politiques plus complexes. S'agissant par exemple des jeux d'argent, nous avons considéré qu'une réflexion sur le poids des outils fiscaux existants et sur les moyens d'accompagner les joueurs excessifs faire primer la création de taxes nouvelles sur les messages publicitaires, assiette qui était du reste assez mal déterminée dans les rédactions proposées. Les amendements relatifs à la taxation des produits sucrés, quant à eux, visaient à retenir des mécanismes tout aussi fragiles et s'exposaient aux observations par nos collègues Chantal Deseyne, Brigitte Devésa et Michelle Meunier dans leur rapport d'information du mois de juin dernier. Mieux vaudrait sans doute recourir prioritairement à l'outil réglementaire pour interdire certaines formes de marketing ou de publicité ou encore fixer des seuils maximaux. En matière fiscale, il serait préférable d'évaluer les outils existants, tels que la taxe sur les sodas de 2018, dont le rapport de bilan est toujours attendu, madame la ministre, et n'en concevoir de nouveaux qu'en donnant un peu de visibilité aux industriels pour reformuler leurs produits.

à certaines des incohérences de la fiscalité sur le tabac en raison de l'inflation. Cette nouvelle contribution, dont l'assiette serait très large, aurait pour conséquence de taxer des produits aujourd'hui exclus intentionnellement de la fiscalité du tabac, comme les cigarettes électroniques traditionnelles.

Monsieur Kern,

des produits du vapotage ». Cette consommation se développe rapidement dans les collèges et les lycées. Parents, directeurs d'établissement scolaire, associations de lutte contre le tabac, s'inquiètent de ce nouveau phénomène de mode, qui peut avoir des conséquences graves.

de mortalité évitable en France. Au cours des dernières années, deux plans pluriannuels ont été mis en oeuvre, mais l'ambition d'une génération sans tabac en 2032 semble rester lettre morte. Selon Santé publique France, plus d'un quart de la population âgée de plus de 18 ans fumait quotidiennement en 2020. de ce phénomène diminue donc insuffisamment et trop lentement, avec ces plans de lutte fondés sur deux piliers : la prévention et la cessation. La politique publique dans ce domaine ne bénéficie que de très peu d'évaluations. À l'occasion des mesures défendues par le Gouvernement dans le cadre de l'article 8,

en a déjà consommé. Pourtant, les risques liés à sa consommation sont nombreux- troubles psychiatriques, états anxio-dépressifs, infarctus -et l'impact est encore plus fort sur les cerveaux en formation, donc sur la jeunesse. C'est d'autant plus inquiétant que la jeunesse française cumule tous les records en la matière : plus d'un tiers des moins de 16 ans ont déjà fumé du cannabis et le taux d'addiction chez nos mineurs est le plus fort d'Europe. Ces statistiques montrent une chose : la politique sanitaire et sécuritaire choisie par la France est un échec. Les sanctions n'ont aucunement endigué la consommation, en particulier chez les plus jeunes.

dans le code des impositions sur les biens et services. Le produit de cette accise sera affecté aux branches maladie, maternité, invalidité et décès du régime général de la sécurité sociale, afin de financer des politiques ambitieuses de prévention et de sensibilisation sur le cannabis. Nous protégerons ainsi la santé psychique et physique des Français. Le cannabis Le cannabis peut et doit être envisagé comme un produit imposable, au même titre que l'alcool ou le tabac. Arrêtons les politiques coûteuses et inefficaces de répression, qui détournent nos forces de l'ordre de missions utiles. Asséchons financièrement les trafics, qui pourrissent le quotidien de certains quartiers. Reprenons la main sur les enjeux de santé publique. Trouvons de nouvelles recettes pour la sécurité sociale. La parole

de la même manière qu'ils boivent de l'alcool ou fument des cigarettes. On peut mépriser davantage les fumeurs de joints que les buveurs de vin, mais ce mépris ne constitue pas une politique publique.

et de lutte contre les addictions.

sur ce sujet, autrement qu'en distinguant entre, d'un côté, les laxistes qui veulent droguer la jeunesse et, de l'autre, les répressifs responsables qui veulent lutter contre le trafic. Je ne connais aucune politique pénale qui soit autant en échec que la politique de lutte contre la consommation de cannabis. Cette politique pénale échoue depuis des années ; elle continue de mobiliser des financements publics importants,

parallèle. D'un point de vue de santé publique, une baisse relative des prix de l'alcool en comparaison des autres produits incite à la surconsommation. Ce phénomène concerne notamment les alcools aux prix déjà faibles et est d'autant plus dangereux qu'il touche encore plus les personnes ayant une consommation excessive, c'est-à-dire 15 % à 20 % de la population de notre pays.

D'autre part, la hausse drastique du prix de l'énergie et des emballages pénalise lourdement les vignerons, qui ne parviennent pas à compenser ces envolées et voient leur chiffre d'affaires diminuer.

ce qui a été dit. Vous savez comme moi qu'un groupe d'experts missionné par Santé publique France a conclu que boire deux verres de vin par jour, et pas tous les jours, n'était pas néfaste à la santé.

À longueur de reportages, sur tous les médias, on nous rappelle les augmentations diverses et variées : +12 % pour ceci, +40 % pour cela ... Nous recevons l'information, mais demeurons dans une sorte de résignation. Daniel Laurent l'a dit, le surcoût des matières premières est une réalité, en viticulture comme ailleurs, que ce soit pour les emballages, les bouchons, les bouteilles, le carburant ... Et je vous fais grâce de celui de l'énergie.

Après l'année noire du covid-19, après les hausses du prix de l'énergie, ce secteur n'a vraiment pas besoin de cela ! Je reprends à mon compte les arguments de Daniel Laurent. Ici, nous ne parlons pas des grands groupes qui sauront amortir les coûts, parlons de petits artisans des TPE, des PME, ancrés dans nos territoires. Contrairement au tabac, il s'agit bien d'une filière agricole- brasseurs, agriculteurs, coopératives, vignerons -ne pouvant accepter ce qui s'apparente à une sanction injustifiée. Cette sanction est d'autant plus injustifiée que cette indexation n'aura aucune aucune conséquence sur la baisse de consommation d'alcool. Bien sûr ! Travaillons plutôt sur la prévention, discutons avec les acteurs du secteur et évitons de stigmatiser une filière déjà lourdement affectée par les crises à répétition. La parole

Le secteur viticole et celui des spiritueux sont des secteurs économiques locaux créant de la richesse et des emplois avant tout dans les territoires ruraux. À ce titre, ils jouent un rôle fondamental pour l'équilibre économique des territoires. L'amendement dont nous débattons vise à déplafonner l'indexation des accises sur l'inflation de la même manière que pour le tabac, alors que les structures des prix de ces produits sont complètement différentes : le tabac est un produit dont le prix est complètement administré par les pouvoirs publics ; l'alcool dépend, lui, d'un prix de marché indépendant de l'État. L'inflation a déjà frappé la filière alcool de plein fouet ces dernières semaines : le prix du verre a grimpé de 60 %, les matières agricoles ont flambé, l'étiquetage a été renchéri. Il n'y a aucune raison d'augmenter encore davantage le prix de l'alcool. De surcroît, nous savons très bien que ce renchérissement se traduira par des importations massives d'alcool depuis l'étranger, dans toutes les zones frontalières de notre pays. « Chers collègues, pour soutenir nos filières et nos emplois, je crois qu'il est important de ne pas porter ce coup de massue à un secteur qui se débat déjà, comme il le peut, avec l'inflation actuelle.

Les trois grands problèmes de santé publique dans notre pays sont le tabac, l'alcool et la pollution de l'air. Madame la ministre, sur le tabac, vous avez baissé le pavillon ; sur l'alcool, vous venez de vous planquer ; sur la pollution de l'air, votre gouvernement a été condamné plusieurs fois. Votre virage de la prévention est à 180 degrés Vous ne traitez aucune des thématiques principales de prévention. Vous vous moquez du monde ! Voilà la réalité, vous ne tenez aucune position courageuse en matière de prévention. Sur lequel de ces trois grands problèmes de santé publique nous proposez-vous d'agir ?

produit légal. Les dommages causés sur l'organisme par la consommation importante de sucre sont connus et documentés : diabète, affections cardiovasculaires, surpoids, cholestérol, hypertension. Le problème de santé publique est réel et doit être traité de manière plus efficace.

Le résultat est sans appel : le volume des ventes de tabac a été divisé par deux entre 1990 et aujourd'hui. Il nous faut employer la même méthode avec les produits les plus sucrés, en premier lieu les sodas. Il existe aujourd'hui une taxe sur le sucre ajouté dans les boissons non alcoolisées, mais son taux est trop faible pour produire de véritables effets en termes de santé publique. Pour la plupart des sodas commercialisés, le montant de la taxe s'élève à moins de 15 centimes par litre de boisson. Nous vous proposons un saut quantitatif qui doublerait le taux de la taxe pour que les prix s'en ressentent et que les habitudes alimentaires en soient modifiées. Nous souhaitons également que la réévaluation soit aussi régulière que pour le tabac, afin de maintenir l'effet dissuasif dans le temps. C'est également un enjeu de finances publiques pour le financement de notre sécurité sociale. La taxe rapporte, dans sa forme actuelle, un peu plus de 480 millions d'euros à la sécurité sociale. Or l'adoption de l'amendement permettrait de doubler cet apport.

Dans ce contexte, il est établi que la consommation de sodas, en particulier chez les plus jeunes, engendre une forte surconsommation de sucre. Il est donc urgent que les pouvoirs publics se saisissent du problème et agissent beaucoup plus fortement contre ce fléau. La taxe soda vise à modifier durablement le comportement du consommateur par la contrainte financière qu'elle fait peser sur lui. L'augmentation substantielle de la fiscalité a une véritable vertu dissuasive et entraîne une baisse importante des achats de boissons sucrées.

Il semblait alors que la taxe soda devait faire l'objet d'une évaluation, notamment dans le cadre d'un comité interministériel pour la santé. Une fois encore, le Parlement ne dispose toujours pas d'informations précises à ce sujet. Cet amendement a pour objet une évaluation sur la mise en oeuvre de la taxe soda adoptée voilà maintenant plus de quatre

ont fait le choix de répercuter intégralement la hausse de la fiscalité sur le prix de vente. Par ailleurs, pour limiter la hausse de prix, certains ont pratiqué une stratégie de réduction de la taille des bouteilles. Ce fameux

qui donnent lieu à des campagnes publicitaires intenses et particulièrement ciblées sur les jeunes publics. Entre 2014 et 2019, les investissements publicitaires des opérateurs de jeux en ligne et paris sportifs ont augmenté de 25 %. D'après les chiffres de l'Autorité nationale des jeux, parieurs sur quatre ont moins de 34 ans. On sait par ailleurs que ce public est particulièrement vulnérable aux phénomènes d'addiction. L'hôpital Marmottan, l'un des principaux centres de soins dédiés à cette question, a observé que les jeunes adultes de moins de 25 ans représentaient à eux seuls 62 % de la totalité des patients pris en charge pour leur addiction aux paris sportifs. En 2019, l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies révélait que les pratiques de jeu à risque modéré ou excessif se retrouvaient plutôt chez les hommes les autres joueurs, issus de milieux modestes et ayant un niveau d'éducation et des revenus inférieurs à ceux des autres joueurs. Grâce au travail de l'ancien Observatoire des jeux- je tiens d'ailleurs à saluer l'implication de Jean-Michel Costes qui fut le premier, dès 2011, à nous alerter sur les dangers de ce phénomène -, il est désormais admis que cette pratique peut entraîner de graves troubles sanitaires et psychiatriques. Devant cet enjeu de santé publique, cet amendement vise à limiter la publicité en ligne afin de réduire l'exposition des plus jeunes, en taxant les investissements publicitaires des opérateurs. La parole Entre 2014 et 2019, les investissements publicitaires des opérateurs de jeux en ligne ont grimpé de 25 %. Les publicités pour les paris sportifs font l'objet de campagnes publicitaires intenses, pendant les compétitions de football, comme ce fut constaté en 2021. Ces publicités aux pratiques contestables poussent aux pratiques excessives. Le résultat est sans appel : dorénavant, 40 % du chiffre d'affaires des opérateurs de jeux d'argent

À propos du poker, celui-ci est associé à la publicité et à la réussite sociale avec des joueurs stars qui gagnent leur vie en jouant et qui sont donc, en quelque

Le nombre de joueurs excessifs a doublé en cinq ans et cela concerne 1,37 million de personnes. L'Autorité nationale des jeux pointe de plus en plus des manquements à l'obligation d'identification et d'accompagnement des personnes dont le jeu est pathologique. nous sommes devant un véritable problème de santé publique : compulsion, dépendance et addiction entraînent en cascade des difficultés sociales, relationnelles, psychologiques et médicales. Ce jeu pathologique est une forme de pratique dans laquelle le joueur perd jusqu'à la notion même du plaisir de jouer. Comme dans toute addiction, il développe une dépendance très forte, il s'engage

Il me semble toutefois que taxer les publicités n'est pas la bonne solution. C'est plutôt en accompagnant ces personnes que l'on réussira le mieux à faire diminuer leur consommation. Par ailleurs, les opérateurs de jeux

pathologies qui sont dues aux substances psychotropes dont nous avons parlé tout à l'heure, comme la cocaïne et l'héroïne. Elle nécessite une thérapie et est donc une source de dépenses de santé. C'est pour cette raison qu'il paraît légitime qu'une taxe contributive des opérateurs de jeux en ligne abonde la branche maladie de la sécurité sociale.

selon Santé publique France. Les entreprises qui incitent à la consommation de cette substance doivent participer à la réduction des effets négatifs liés à l'alcool. C'est pourquoi cet amendement vise à soumettre les alcooliers à une taxe sur la publicité pour les produits alcooliques. Le produit de la taxe, soit 25 millions d'euros, sera dédié à la prévention des dommages liés à la consommation d'alcool. L'alcoolisme est un fléau. Les personnes qui sont touchées peuvent vivre un calvaire et un enfer toute leur vie et le faire vivre également à tout leur entourage, particulièrement aux enfants. Constituant une source de recettes fiables, cette taxe permettra de concrétiser l'engagement pris par le Gouvernement au travers de la stratégie décennale de lutte contre les cancers 2021-2030 : faire de la prévention une priorité de la politique de santé publique.

Des données incontestables montrent que la commercialisation d'aliments nocifs pour la santé et de boissons sucrées a un lien avec l'obésité de l'enfant. Même si l'industrie déploie un nombre croissant d'initiatives volontaires, l'exposition à la commercialisation des aliments nocifs pour la santé reste un problème majeur, appelant un changement pour protéger tous les enfants de façon égale. Le packaging, les publicités colorées, gaies et alléchantes ont des effets non négligeables sur les enfants. En l'absence de cadre contraignant, cet amendement vise à soumettre la publicité en faveur de ces produits, c'est-à-dire de l'alimentation ultratransformée, au versement d'une contribution dont le produit sera affecté à la branche maladie de la sécurité sociale dans un but de prévention.

prescripteurs de comportements délétères et surfant sur des modèles consuméristes. Et je vous parle d'une alimentation n'ayant rien à voir avec ce que l'on entend traditionnellement par-là : elle est issue d'un mélange de briques alimentaires, d'arômes artificiels, d'exhausteurs de goût,

nutritionnel. Le marketing alimentaire à destination des enfants et des adolescents fait malheureusement la promotion de denrées alimentaires à faible intérêt nutritionnel. Il est avéré qu'une surconsommation d'aliments industriels, notamment de produits ultratransformés, favorise la survenance de pathologies chroniques- nous en avons parlé.

Cet amendement vise à instaurer le versement d'une contribution au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie par les annonceurs et promoteurs de tout type de messages publicitaires et de promotions à l'intention des enfants et adolescents pour des denrées alimentaires défavorables pour la santé. L'étiquetage nutritionnel obligatoire et le Nutri-score permettent d'évaluer la composition de ces produits et leurs conséquences défavorables pour la santé. Les compétences techniques

des organismes complémentaires à un taux de 0,8 % sur une assiette similaire à celle de la taxe de solidarité additionnelle, pour un rendement proche de 300 millions d'euros. L'idée d'un partage entre les régimes de base et les organismes complémentaires

Pour notre part, nous sommes particulièrement attachés au financement de la sécurité sociale par les cotisations sociales. La pédagogie étant l'art de la répétition, je le redis encore une fois : nous rejetons la fiscalisation de la sécurité sociale. Pour nous, cette dernière doit rembourser intégralement les dépenses de santé sans reste à charge pour les assurés sociaux. Les organismes complémentaires doivent se concentrer sur leurs missions de prévention et de gestion des établissements de santé, ainsi que des résidences pour personnes âgées. C'est la raison pour laquelle nous sommes opposés à la mise à contribution des organismes complémentaires à la sécurité sociale, d'autant que, en l'état de la rédaction de l'article et des amendements proposés, ce sont les adhérents des complémentaires

Pour toutes ces raisons, nous voterons contre les amendements proposés en ce sens, notamment

Cette pratique permet aux complémentaires santé de moins bien rembourser leurs assurés qui ne se rendraient pas chez un professionnel de santé affilié à leur réseau de soins, y compris lorsque celui-ci est leur professionnel de santé habituel. Le niveau de remboursement des assurés peut varier du simple au double chez certaines complémentaires mesure où de nombreux territoires ne disposent pas de professionnels de santé affiliés à ces réseaux, le remboursement différencié peut également aggraver les inégalités territoriales d'accès aux soins. Par ailleurs, cette pratique va à l'encontre des objectifs fixés par le « 100 % santé », puisqu'elle complexifie la lisibilité des droits et garanties auxquels les assurés peuvent prétendre. Enfin, elle rompt le caractère solidaire du contrat responsable. C'est pourquoi il est proposé de subordonner les avantages fiscaux accordés aux complémentaires santé à une modération de l'ampleur de la différenciation des remboursements.

Pour être qualifiés de responsables, les contrats des complémentaires santé doivent couvrir non seulement le ticket modérateur, mais également les paniers « 100 % santé » en optique, en dentaire, en audiologie, quel que soit le professionnel auquel l'assuré s'adresse. Il ne peut donc pas y avoir de remboursement différencié sur ces équipements, que ceux-ci aient été achetés dans un réseau de soins

prenant en charge l'activité physique ou des séances de diététique, par exemple. Dans ce cadre, il est précisé que les mutuelles ne recueilleront pas d'informations médicales auprès de l'assuré ou des personnes souhaitant bénéficier de cette